La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du mercredi 17 juin a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire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

afin de limiter la circulation des documents, vous êtes invités à utiliser vos tablettes et la fonctionnalité « En séance » sur notre site internet pour prendre connaissance du dérouleur et des amendements. Des liasses resteront à votre disposition, à la demande.

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, au mois de mars dernier, une situation exceptionnelle a justifié l'instauration d'un régime exceptionnel. Il le fallait, et nul ne pense aujourd'hui que cet état d'urgence sanitaire était au mieux une option regrettable, au pire une fantaisie catastrophiste. Il l'était d'autant moins qu'il a été scrupuleusement travaillé, amendé, enrichi par les représentants de la Nation, car, quelles quelles que soient les épreuves que nous traversons, notre arme la plus efficace demeure la démocratie. L'état d'urgence sanitaire expirera le 10 juillet prochain. La fin de l'état d'urgence signifie-t-elle la fin de l'épidémie ? J'aimerais vous dire que oui. J'aimerais vous dire que le pire est derrière nous et que nous pouvons sans crainte retrouver une vie qui soit sereine, à défaut d'être insouciante ... Mais ce serait malheureusement ce serait malheureusement irresponsable. Les indicateurs sont certes rassurants, mais nous devons tous rester vigilants. Le Gouvernement ne demandera pas une seconde prolongation de l'état d'urgence sanitaire, qui prendra donc fin comme prévu le 11 juillet prochain. La sortie de l'état d'urgence doit toutefois être organisée, parce que la prudence reste de mise et que de nombreuses mesures garderont toute leur pertinence dans les mois à venir. Le choix éthique que nous devons faire est celui de la responsabilité. de l'état d'urgence sanitaire n'est plus justifiée, il ne faut pas nous bercer d'illusions et faire comme si les risques de redémarrage de l'épidémie n'existaient pas. Ces risques existent bel et bien, et une sortie précipitée de l'état d'urgence sanitaire ne ferait qu'augmenter leur poids. Les deux articles de ce projet de loi ont fait l'objet de débats nourris à l'Assemblée nationale, qui a adopté plusieurs modifications. La durée modifications. La durée du régime transitoire, initialement prévu jusqu'au 10 novembre, a été raccourcie au 30 octobre. Par ailleurs, ce régime transitoire conserve des mesures dont la pertinence est indiscutable, y compris pour ceux qui ne sont pas épidémiologistes- nous sommes encore nombreux dans ce cas

Ces trois items ont fait l'objet de débats en commission ce matin, et nous aurons de nouveau des échanges sur ces sujets lors de l'examen des articles ce soir. L'application de la plupart des autres mesures prévues pendant l'état d'urgence sanitaire restera possible, mais dans les conditions du droit commun du code de la santé publique ou du code de commerce,

L'ensemble du dispositif devra en tout état de cause être réexaminé, puisque vous avez prévu qu'il deviendra caduc à compter du 1 avril 2021. Il faudra alors le repenser ensemble, à la lumière de l'expérience acquise, en espérant de tout coeur que ce virus aura alors trouvé sa place dans les livres d'histoire et qu'il aura complètement disparu de notre quotidien. Mesdames, messieurs les sénateurs, la sortie de l'état d'urgence que nous construisons dans ce projet de loi n'est pas une sortie sèche, parce que nous ne voulons pas faire comme si nous étions définitivement à l'abri du risque épidémique. Rien ne serait pire que la précipitation : ce serait tout à la fois oublier bien vite les semaines terribles que nous venons de connaître et augmenter le risque d'en connaître à nouveau. Je crois d'ailleurs que les Français sont sensibles à ce point.

L'état d'urgence sanitaire a été voté dans cet hémicycle, et je sais que vous vous êtes toujours montrés, à juste titre, très vigilants et exigeants. L'état d'urgence sanitaire a eu des conséquences lourdes, très lourdes, notamment Le Président de la République n'a pas manqué de rappeler que nous avions fait passer la santé avant le reste, « quoi qu'il en coûte ». Si c'était à refaire, nous ne ferions pas autre chose,

L'utilité de prolonger la durée de conservation des données pseudonymisées pour la recherche et la veille épidémiologiques est bien réelle. Mesdames, messieurs les sénateurs, si nous avions quelques points de désaccord, je reconnais et salue le travail constructif de la commission et vous remercie de donner au Gouvernement les moyens d'agir pendant cette phase nouvelle de gestion de la crise qui s'ouvrira à compter du 11 juillet prochain. La santé de nos concitoyens

Monsieur le président, je suis très heureux de retrouver cette tribune, qui nous a manqué au cours des derniers mois Monsieur le ministre, je vous remercie des explications que vous nous avez apportées. Mes chers collègues, je suis heureux de vous retrouver pour ce débat très important. Monsieur le ministre, la commission des lois s'est réunie ce matin. Nous travaillons dans des conditions extrêmement tendues. Nous avons déjà accepté de le faire pour faire aboutir la loi du 23 mars dernier, puis celle du 11 mai dernier. Nous espérions que la sortie de l'état d'urgence sanitaire justifierait que le Parlement dispose de davantage de temps

Nous avons décidé de substituer à l'article 1 des dispositions qui nous semblent exactement proportionnées à vos besoins. Il vous reviendra de nous dire si nous y sommes parvenus, car il faut naturellement que vous puissiez amener progressivement à la sortie de l'état d'urgence en disposant des moyens qui vous seront nécessaires. Il n'est pas question pour nous de vous les marchander. Nous tenons simplement à vous rappeler que, en matière de libertés essentielles, il n'y a aucune raison que le législateur vous autorise à faire plus que ce qui vous semble à vous-même nécessaire et que nous pourrions approuver après discussion avec vous. Cette discussion n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière en commission compte tenu de votre emploi du temps

reconduction, tout en vous rappelant que si les conditions qui justifient l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en Guyane devaient fort heureusement disparaître, rien ne vous imposerait alors de maintenir cet état d'urgence sanitaire localement pendant les quatre mois

protecteur. Nous avons eu une discussion assez longue sur votre souhait de prolonger les durées de conservation des données recueillies dans le cadre des systèmes d'information pour le dépistage

de sortie de l'état d'urgence, mais un texte de prorogation des principales mesures de l'état d'urgence. Si le Sénat est suivi, ce sera un texte de sortie de l'état d'urgence. Nous sommes allés jusqu'à modifier le fameux article L. 3131-1

C'est pourquoi nous avons bien précisé que vous pouvez à tout moment prendre un décret pour déclarer l'état d'urgence sanitaire et prendre toutes les mesures auxquelles nous avons consenti au mois de mars dernier dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, oui à la vigilance, nous avez-vous dit, monsieur le ministre, mais non à l'état d'urgence. Nous avons bien compris votre approche et votre raisonnement.

J'ai parfois l'impression que certains de nos compatriotes dorment sur un volcan : tout semble aller bien, mais vous savez que le virus peut toujours se réveiller.

Notre collègue député Hervé Saulignac l'a dit à l'Assemblée nationale : vous créez quelque chose de neuf. On connaissait le droit commun, on connaissait l'état d'urgence, et vous créez une sorte de pseudo-état d'urgence à géométrie variable et à durée aléatoire, donc quelque chose de bizarre.

Par prudence, nous avions également déposé des amendements de repli, l'un pour garantir la liberté de circulation- sur ce point, M. Bas est allé à notre rencontre ou nous sommes allés à la sienne, peu importe

rénové. Notre position est à cet égard très claire. J'ajoute quelques mots pour nos collègues de l'outre-mer et, tout particulièrement, pour Mme Catherine Conconne, qui, au nom de plusieurs de ses collègues,

-en toute sérénité dans leurs territoires. De même, il nous paraît nécessaire que des mesures spécifiques soient prises s'agissant de Mayotte et, surtout, de la Guyane.

qui se réduirait à cet article. En effet, je dois dire que, à mon sens- je rejoins ainsi les propos de M. Bonnecarrère -, l'Assemblée nationale a fait un bon travail. Il me semble que, dès lors que le recueil des données est prolongé pour une durée très limitée et exclusivement pour des impératifs de recherche scientifique, il est raisonnable et peut être approuvé. Voilà les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous pensons que ce texte n'est pas utile sous cette forme

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, à l'heure où nous parlons, la vie des Français poursuit son retour vers la normalité et, avec elle, l'application des lois de la République. Une grande part de l'activité économique a repris, avec, dès la première heure ce matin, la réouverture des cinémas, des centres de vacances et des casinos. Le retour en classe signe également la reprise de l'école républicaine obligatoire. C'est aussi, pour tous les élèves concernés, un moyen de retrouver camarades et professeurs pour clore symboliquement l'année scolaire avant les grandes vacances, après l'expérience souvent difficile du confinement. Hier, déjà, dans les villes où elle n'avait pas été interdite, la fête de la musique a pu être célébrée, parfois avec des débordements, mais toujours dans un grand élan de liberté retrouvée, après des mois d'isolement. âgées dépendantes (Ehpad), la situation sanitaire est désormais sous contrôle, à l'exception de certains territoires français d'outre-mer- je pense à Mayotte et à la Guyane où la situation est toujours préoccupante, j'y reviendrai. Dans quelques jours, nos concitoyens seront également appelés à voter pour le second tour des élections municipales, après une période inédite de suspension de la vie démocratique locale. Tous ces éléments laissent à penser que l'urgence sanitaire est dernière nous. Si tel est le cas, le maintien de l'état d'urgence n'est plus justifié. Devant les juridictions, le retour à la normale ne manque pas de fragiliser les actes et les décisions pris sur le fondement de l'état d'urgence sanitaire. Le 13 juin dernier, par exemple, une ordonnance de référé du Conseil d'État a suspendu la décision d'interdiction des manifestations organisées par l'association SOS Racisme et plusieurs syndicats. Après les nombreux bouleversements que nous venons de connaître, il importe que les règles applicables soient claires et les plus stables possible, afin de ne pas ajouter aux déstabilisations qui minent déjà le pays. Le retour au droit commun doit être la norme. Au moment de la prorogation, nous avions insisté sur l'importance du principe de proportionnalité des mesures prises par rapport aux circonstances de temps et de lieu. Certains juristes regrettaient d'ailleurs que ce principe n'ait pas été appliqué plus rigoureusement dans les zones épargnées par le virus au nom de la protection des libertés. La lecture des dispositions du code de la santé publique par le Conseil d'État est dorénavant claire : il en résulte que, sous le régime de l'état d'urgence sanitaire, les manifestations et les rassemblements ne sont illégaux que si les circonstances épidémiques le justifient et aucune précaution sanitaire adaptée n'est prise. Nous aborderons l'examen de ce texte avec ce même souci de la protection des libertés. Or l'article 1 du projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui permet au Premier ministre, en même temps qu'il met fin à l'état d'urgence en France métropolitaine et dans la plupart des territoires d'outre-mer,

à l'heure actuelle, il n'existe pas de consensus scientifique, tant ce virus demeure mystérieux. Toutefois, les dernières semaines nous permettent d'exercer une vigilance optimiste, comme au moment de la prorogation de l'état d'urgence, dont la durée avait d'ailleurs été raccourcie du 23 juillet au 10 juillet par le Sénat, une position défendue par notre collègue Joël Labbé et plusieurs membres du groupe du RDSE. Nous étions donc majoritaires

des amendements votés à l'Assemblée nationale et de ceux qui ont été adoptés ce matin sur l'initiative de notre rapporteur, la majorité d'entre nous s'apprêtent désormais à se prononcer en sa faveur, en vue d'une sortie définitive à l'automne. L'article 1 en ressort quasiment vidé de sa substance initiale. En définitive, nos réserves portent essentiellement sur la façon de légiférer. Cette période a considérablement affaibli l'autorité de la loi, soit en la marginalisant au profit des ordonnances,

Il n'était pas très respectueux du Parlement de mettre une nouvelle fois ce sujet sur la table, comme l'article 2 du projet de loi le prévoyait avant l'intervention des deux chambres. Lorsque la crise sera véritablement derrière nous,

il eût été préférable, disait-il, « de légiférer à ce sujet de manière abstraite et générale, c'est-à-dire de faire une loi en une période où elle n'aurait pas eu à s'appliquer dans l'immédiat et de ne pas prendre le prétexte d'une situation spéciale et contemporaine sur un point du territoire pour provoquer une intervention législative Ses mots restent d'actualité. N'oublions pas, enfin, la situation des outre-mer et les efforts que continuent de fournir ceux de nos concitoyens qui se trouvent aux confins du territoire français. Ce n'est en réalité que le début de la fin de l'état d'urgence, pour reprendre le nom initial du projet de loi. Alors que le virus continue de circuler, cette vigilance optimiste que j'évoquais reste de mise. Aujourd'hui, elle passe essentiellement par le respect des gestes de précaution que chacun d'entre nous connaît désormais.

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Alors que l'état d'urgence a été prorogé jusqu'au 10 juillet, il est nécessaire de créer toutes les conditions favorables à la confirmation, dans les semaines et les mois à venir, de l'amélioration de la situation sanitaire de notre pays. Pour ce faire, le texte

Il me semble que le Gouvernement, la majorité à l'Assemblée nationale et la commission, ce matin, par la voix du rapporteur, ont plutôt répondu favorablement à la première question : oui, nous avons encore besoin de mesures spécifiques. Certes, la situation s'améliore,

plus aucune mesure ne se justifie. Il faut choisir parmi les critiques : à partir du moment où la situation n'est pas entièrement stabilisée, une sortie sèche

pourra être conclusive sur ce point à l'issue des débats. Au terme de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale et en commission, nous pouvons affirmer qu'il ne s'agit pas d'un état d'urgence déguisé, qui tairait son nom en vertu d'une pudeur mal venue. Si les deux régimes peuvent se ressembler, c'est aussi par les garanties le caractère proportionné, approprié et nécessaire des mesures prises, toujours sous contrôle du juge administratif, qui peut être saisi en référé. Je pense aussi à la faculté de contrôle et d'évaluation du Parlement sur les mesures prises, ce qui permet d'envisager

sur la situation en Guyane : au regard de l'évolution de l'épidémie et du pic qui est attendu, il n'est pas possible de ne pas soutenir la prorogation de l'état d'urgence. Sur la situation spécifique de Mayotte,

Le Gouvernement a décidé de ne pas prolonger officiellement l'état d'urgence sanitaire, qui devait prendre fin le 10 juillet, mais d'organiser une période dite « transitoire », qui permettra au Premier ministre, durant les trois mois et demi qui suivront la fin de l'état d'urgence, de réactiver par voie de décret plusieurs dispositions déployées dans le cadre même de cet état d'exception. Autrement dit, au lieu de solliciter l'avis du Parlement pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, le Gouvernement lui demande de lui octroyer, d'un coup, toutes les compétences- ou presque -utiles pour agir seul par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne les déplacements et l'accès aux transports, l'ouverture des établissements recevant du public et les rassemblements sur la voie publique. font dire à Stéphanie Hennette-Vauchez, professeure de droit public, qu'il s'agit là « d'enrichir la grammaire des droits d'exception d'un nouveau régime dérogatoire ». En plus du droit commun et de l'état d'exception, il y aurait désormais la « sortie une sorte de zone grise dans laquelle on ne sait pas vraiment si l'on est dans ou en dehors de l'état d'urgence. Néanmoins, pourquoi vouloir mettre en place un tel régime ? Selon nous, celui-ci est profondément inutile, tant le Gouvernement dispose déjà de tous les outils pour faire face à une nouvelle situation de crise : comme certains l'ont déjà dit, l'article L. 3131-1 du code de la santé publique offre déjà des pouvoirs extrêmement larges au ministre de la santé en cas de circonstances exceptionnelles. Un décret pour les réactiver aurait suffi en cas de deuxième vague. Nous le savons, le risque zéro n'existe pas, et plusieurs foyers endémiques resurgissent sur la planète. Mais n'avez-vous pas toutes les compétences nécessaires en cas de résurgence du virus dans notre pays ? N'êtes-vous pas prêt à y faire face normalement, en ayant recours au droit commun, comme le font d'ailleurs les pays européens voisins ? Ne devriez-vous pas plutôt continuer à consolider notre système de soins et à combler les carences en personnel au lieu de rogner sur nos libertés publiques ? aide alimentaire, précarité énergétique, moratoire sur les loyers, gratuité des transports en commun pour les travailleurs, toute une série de mesures sociales auraient eu leur place dans un tel texte pour une réelle sortie de l'état d'urgence humaine et efficace, qui réponde aux préoccupations des Français et les rassure. L'heure est davantage à l'état d'urgence social qu'au prolongement d'un état d'urgence coercitif. Pourquoi décider de sortir de l'état d'urgence dans ces conditions ? C'est presque pire qu'une simple prolongation ! On nous demande de ne conserver que les mesures restrictives de liberté, alors qu'il existe des mesures pour faire face à une nouvelle crise. Les peurs légitimes qu'a engendrées la crise sont ici instrumentalisées pour confiner nos libertés. Comme « avoir peur, Comme « avoir peur, c'est se préparer à obéir », pour reprendre les mots de Hobbes, il est bien connu que la peur est un outil aisé à mobiliser pour des politiques requérant une adhésion aveugle.

quelles qu'elles soient, policières ou sociales. Nous vivrons encore avec ce virus, ou avec d'autres : alors, l'exception ne sera plus, et les dispositions deviendront communes. Nous définissons aujourd'hui les conditions dans lesquelles nous souhaitons gérer les urgences sanitaires nous ne voulons certainement pas le faire en limitant nos libertés publiques, pas plus qu'en étendant les méthodes de surveillance généralisée et le stockage des données personnelles, comme le propose l'une des mesures de ce projet de loi. Quoi que vous puissiez en dire, les risques de marchandisation des données sont réels, sans parler des ressources et du budget que tout cela nécessite. Quant à l'application StopCovid, c'est un fiasco, puisqu'elle n'a été activée que par 2 % de la population et que le nombre d'utilisateurs actifs est évalué par des chercheurs- pas par moi ! -à 0,5 % de la population française

que le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. Finalement, vous l'aurez bien sûr compris, nous nous opposerons à ce texte. Certes, la commission des lois propose de réglementer plutôt que d'interdire, mais avouons resterions ainsi au milieu du gué. Sur le fond, ce projet de loi est inutile, parce qu'il met en place un régime d'exception hybride et dangereux, en pérennisant des mesures qui portent atteinte à notre droit commun. Et cela, j'en suis désolée, monsieur le ministre, mais nous n'en voulons pas

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l'épidémie semble sous contrôle pratiquement partout sur le territoire métropolitain. L'État doit néanmoins continuer à accompagner les territoires dans lesquels le virus circule encore très activement,

La crise sanitaire, que nous espérons être derrière nous, a coûté la vie à près de 30 000 de nos compatriotes. Ce virus a beaucoup perturbé la vie de nos concitoyens,

moins importantes, notamment en raison du contexte social tendu dans lequel notre pays est plongé depuis plusieurs mois. C'est le cas de la possibilité de restreindre la liberté de manifester. Dès la fin du confinement, en dépit des interdictions,

la possibilité de réglementer ces rassemblements. L'exercice n'est pas simple, et il est particulièrement sensible ! Ainsi, le texte prévoit de soumettre les manifestations sur la voie publique à autorisation, eu égard à la mise en oeuvre des mesures barrières destinées à lutter contre l'épidémie.

Il en sera de même pour la restriction de la liberté d'aller et venir des individus ou encore la réglementation de l'ouverture des établissements recevant du public. Ces mesures sont fortement attentatoires aux libertés individuelles. Nous devons donc veiller à ce qu'elles répondent à des circonstances très précises et qu'elles soient aussi limitées que possible dans le temps. Force est de constater qu'elles ne seront pas nécessaires partout, car tous les territoires de la République n'ont pas été touchés de la même manière par le virus- certains ont eu la chance d'être plus épargnés que d'autres. De ce fait, il nous semble important, dans une logique de décentralisation, que le partage de compétences entre l'État et les collectivités locales soit clarifié, en particulier dans les territoires ultramarins. Les collectivités doivent avoir les moyens de protéger au mieux leur population.

Les mesures barrières devront être appliquées tant que le virus n'aura pas disparu et qu'un traitement ne sera pas disponible. La période qui s'ouvre sera déterminante. La résurgence du virus dans plusieurs pays doit nous inciter à la prudence le groupe Les Indépendants soutient les objectifs portés par ce projet de loi : il nous faut sortir de l'état d'urgence, tout en restant sur nos gardes. Mais les mesures prises pour faire face à cette situation exceptionnelle

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, chers collègues, ce texte s'inscrit dans la droite ligne des deux lois que nous avons précédemment votées dans le cadre de cette épidémie de Covid-19 : la loi du 23 mars 2020 et la loi du 11 mai 2020. Ces deux textes avaient notamment pour objet de donner au Gouvernement des prérogatives lui permettant de prendre des mesures adaptées à la gravité de la situation sanitaire que nous connaissions, en raison de la

prenait acte d'une amélioration de la situation sanitaire et facilitait ce que l'on a appelé le « déconfinement », c'est-à-dire le desserrement progressif des restrictions appliquées à notre vie quotidienne.

Pour respecter les principes de nécessité et de proportionnalité fixés par le législateur pour recourir à l'état d'urgence sanitaire, le moment est venu d'ouvrir un nouveau cycle dans la gestion de l'épidémie de Covid-19, qui permette tout à la fois de répondre à l'aspiration collective au rétablissement du droit commun et de garder la capacité d'agir rapidement face à une éventuelle dégradation de la situation sanitaire, à plus forte raison pendant la période estivale ». J'avoue que je n'enlèverai pas une virgule à cette phrase ! C'est exactement ce que l'on souhaite faire au travers de ce texte, et c'est, me semble-t-il, parfaitement

en oeuvre ce que décrivait le Gouvernement dans son exposé des motifs, c'est-à-dire une sortie graduelle de l'état d'urgence, au travers de mesures certes nécessaires, mais aussi proportionnées à l'état sanitaire du pays,

est-il inscrit dans la position de la commission des lois ? Tout d'abord, en lieu et place des interdictions, nous nous contentons de réglementations, ce qui est tout de même sensiblement différent, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Ensuite, nous rétablissons le principe de la liberté, qui doit rester le principe en droit français,